de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Cet échange fructueux s'est également noué au stade de la ratification de l'ordonnance, tant dans cet hémicycle que dans celui du Palais-Bourbon. Le Gouvernement salue à cet égard le travail accompli par le rapporteur de votre commission des lois, François Pillet, qui a su mener une analyse précise des dispositions de l'ordonnance pour en améliorer certains points, tout en faisant preuve d'un grand esprit d'ouverture et de responsabilité. En effet, première assemblée saisie de ce texte, le Sénat, sur l'initiative de son rapporteur, a opportunément clarifié le sens de certaines dispositions de l'ordonnance, sans toutefois en modifier l'esprit. L'Assemblée nationale, de la même manière, n'a pas remis en cause certaines de ces améliorations et n'a apporté que de rares, mais utiles, nouvelles modifications, de sorte que de nombreux points ne sont plus, aujourd'hui, en débat. Ainsi en est-il de la consécration de la jurisprudence, qui exclut du champ de la réticence dolosive l'estimation de la valeur de la prestation, des règles relatives à la capacité des personnes morales ou aux conflits d'intérêts en matière de représentation ou encore de la définition du préjudice réparable en cas de rupture fautive des négociations. au-delà des améliorations apportées au texte même de l'ordonnance, votre commission des lois, par ses travaux nourris, a dégagé en première lecture des lignes d'interprétation claires, notamment sur les questions d'articulation entre le droit commun et les droits spéciaux

pour les praticiens, qui disposeront ainsi de travaux préparatoires enrichis. Cette deuxième lecture s'ouvre donc, grâce à ce dialogue des chambres marqué par la volonté de tendre vers le compromis, sur un texte amélioré, dont l'équilibre et l'esprit restent fidèles à ceux que le Gouvernement a entendu lui conférer : concilier l'efficacité économique du droit et le renforcement de la justice contractuelle.

il s'agit des prérogatives du juge en matière d'imprévision. En effet, alors que l'ordonnance a enfin doté le droit français d'un mécanisme permettant de prendre en compte un changement de circonstances imprévisible venu bouleverser l'économie du contrat et de restaurer l'équilibre initialement voulu par les parties, votre commission propose de revenir sur ce texte et de limiter les pouvoirs du juge saisi par une seule des parties à la seule résolution résolution du contrat, excluant ainsi la possibilité pour le juge, saisi par une seule des parties, de réviser ce contrat. Les objections du Sénat sont connues. Elles tiennent principalement à l'atteinte qui serait portée à la force obligatoire du contrat et à la liberté contractuelle. Le Gouvernement les avait bien évidemment à l'esprit. C'est d'ailleurs précisément pour ne pas porter à ces principes essentiels du droit des contrats une atteinte injustifiée que la possibilité ouverte par le dispositif instauré par l'ordonnance a été strictement encadrée, ainsi que j'aurai l'occasion de le rappeler lors de l'examen de l'amendement déposé par le Gouvernement. L'incidence négative sur l'attractivité du droit français a également pu être mise en avant. Le renforcement de l'attractivité de notre droit est précisément l'un des objectifs de l'ordonnance. À cet égard, le Gouvernement a rappelé que cette disposition était supplétive, que les parties pouvaient choisir de l'écarter et que son incidence ne serait donc que limitée dans les contrats internationaux. Le Gouvernement estime surtout que la modification proposée par votre commission ôte à ce dispositif novateur son utilité et son efficacité. En effet, il est très peu probable que des parties qui ne se seraient pas accordées sur les termes de la renégociation, voire sur la nécessité même de renégocier, décident finalement de s'accorder pour confier ce pouvoir au juge. Le Gouvernement estime qu'il peut justement être de l'intérêt des parties de permettre au juge, dans certaines circonstances, de « laisser une dernière chance » au contrat. Il ne s'agit pas de donner au juge le pouvoir de faire le contrat, mais de l'adapter, en restaurant les équilibres initialement voulus par les parties que leurs désaccords passés ne leur permettent plus de rétablir par elles-mêmes. S'il est évident qu'il doit pouvoir être mis fin à une relation contractuelle dont le maintien à tout prix est contraire à l'intérêt des parties, il est toutefois des cas dans lesquels la résolution du contrat ne présente, ne présente, à l'inverse, d'intérêt économique pour aucune des parties, par exemple si des emplois devaient être menacés par la fin du contrat en question. C'est précisément pour cela que le juge doit, à notre sens, disposer d'une option et pouvoir, selon les circonstances, maintenir le contrat, en restaurant l'équilibre initialement voulu par les parties. Notre tradition juridique a tendance à favoriser la survie du contrat. Permettre aux parties, puis au juge, en cas d'échec des négociations, de la favoriser ou, si les circonstances le justifient, d'y mettre fin ne fait qu'adapter cette tradition aux évolutions économiques susceptibles d'affecter les situations contractuelles. Il ne s'agit nullement de favoriser un quelconque interventionnisme judiciaire. D'une manière générale, l'ordonnance privilégie, notamment en cas d'inexécution du contrat, des mécanismes extrajudiciaires : résolution unilatérale, réduction du prix ... Cela évite aux parties le temps et le coût d'une procédure judiciaire. Cependant, l'intervention du juge paraît indispensable lorsqu'il faut concilier la force obligatoire du contrat et une certaine forme de justice contractuelle. Votre assemblée l'a d'ailleurs bien compris, en confirmant la pertinence de l'introduction d'un mécanisme judiciaire de révision pour imprévision. Le Gouvernement propose simplement d'aller plus loin et estime qu'il serait regrettable de ne pas donner au juge une autre option que la fin du contrat. De la même manière que le maintien de la relation contractuelle n'est pas toujours la solution idéale, sa rupture n'est pas toujours la solution économiquement la plus adaptée. Le Gouvernement est donc très attaché à ce que cette disposition emblématique et novatrice de l'ordonnance soit maintenue et que sa pleine efficacité lui soit restituée, afin de conserver à l'ordonnance l'équilibre auquel elle était, de l'avis général, parvenue. illustrerait parfaitement la qualité des échanges, dont la présente ratification a été l'occasion, ce dont, au nom du Gouvernement, je vous remercie.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons en nouvelle lecture le projet de loi devant nous amener à ratifier l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, déjà entrée en vigueur le 1 octobre 2016, soit il y a seize mois. Bien qu'ayant été, depuis l'origine, opposé à l'utilisation d'une ordonnance pour effectuer une réforme sur plus de 300 articles du code civil, animée par des choix politiques et ne portant pas seulement sur des aménagements techniques, le Sénat, dans un esprit de responsabilité, a choisi de ne pas engager « la réforme de la réforme ». Lors des débats devant l'Assemblée nationale, vous avez indiqué, madame la garde des sceaux, que « le Sénat avait fait preuve de responsabilité en n'apportant au texte de l'ordonnance que de rares modifications au regard de son ampleur et et en permettant, par les débats qui s'y sont déroulés, de résoudre d'éventuelles difficultés d'interprétation ». Vous venez de confirmer ce propos et je vous en remercie. Toutefois, il n'est pas satisfaisant de devoir ratifier l'ordonnance après presque un an et demi d'application des dispositions qu'elle contient, alors même que quasiment huit mois se sont écoulés entre sa publication et son entrée en vigueur. La prochaine révision constitutionnelle nous permettra certainement d'interdire, à l'avenir, ce genre de situation, ... Certainement ... ... dont chacun admettra le caractère potentiellement néfaste sur la stabilité du droit. Sur le fond, je reconnais que le travail accompli au sein de notre assemblée a été largement respecté par nos collègues députés, par ailleurs tenus d'examiner ce texte dans des délais très contraints. Ils se sont limités, pour l'essentiel, à examiner les modifications issues des travaux du Sénat, en n'abordant qu'un seul sujet nouveau- au demeurant utile, technique et circonscrit -, qui concernait le sort des sûretés en cas de cession de contrat et de cession de dette.

La commission des lois vous propose de retenir certaines modifications effectuées par l'Assemblée nationale et d'adopter des rédactions de compromis raisonnables par rapport à celles qui ont été adoptées en première lecture. Madame la garde des sceaux, vous avez considéré devant l'Assemblée nationale que « le Sénat a contribué à clarifier le texte de l'ordonnance, sans en modifier ni le sens ni l'esprit ». Vous avez aussi salué le « dialogue fructueux qui s'est noué depuis le début du processus de ratification ». Je relève que ce fut encore le cas dans la poursuite du dialogue avec les représentants du ministère de la justice dans le cadre de cette seconde lecture, où nous sommes ensemble restés attentifs aux commentaires publiés par la doctrine ces dernières semaines, ainsi qu'aux travaux menés par nos deux assemblées Ainsi, sur la définition du contrat d'adhésion, laquelle conditionne la possibilité de contester le caractère abusif de certaines clauses du contrat devant le juge, le Gouvernement avait partagé l'analyse du Sénat en première lecture, ce qui ne fut pas le cas de nos collègues députés. En parfait accord entre nous, le Gouvernement a donc présenté en commission une rédaction améliorée, très proche de la rédaction du Sénat de première lecture, que nous avons pleinement approuvée. uniquement deux points de désaccord, qui sont d'inégale importance. Tout d'abord, les dispositions relatives à la révision judiciaire pour imprévision, qui portent, à notre avis, une atteinte disproportionnée au principe de de la force obligatoire du contrat et altèrent gravement l'image du droit français. Ensuite, les dispositions relatives à l'application de la réforme aux contrats antérieurs, qui doivent exprimer clairement la volonté- au demeurant

pourrait apparaître comme une révolution, monsieur le rapporteur, mais n'en est pas réellement une. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'aurait pas accepté d'assumer ce risque, il peut y avoir renégociation du contrat.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le Sénat tout entier s'était opposé, en 2015, à ce que le Gouvernement procédât par ordonnance à la réforme la plus ambitieuse du code civil depuis 1804. Il y a plus d'un an, le 1 octobre 2016, l'ordonnance est entrée en vigueur. Lors des travaux en commission, il est apparu particulièrement important de ne pas créer un droit intermédiaire, qui ne s'appliquerait qu'aux contrats passés entre octobre 2016 et la promulgation de la loi de ratification, afin d'éviter de faire coexister trois régimes juridiques simultanément. C'est pourquoi le rapporteur, François Pillet, dans un esprit de responsabilité, a estimé qu'il fallait ratifier l'ordonnance sans modifications majeures. Cette réforme de grande ampleur du droit des contrats, du régime général des obligations et du régime de la preuve des obligations est nécessaire et attendue. Elle paraît largement approuvée. Renforcer la sécurité juridique et l'attractivité du droit des contrats, le moderniser, le rendre plus lisible sans le bouleverser, l'adapter aux enjeux contemporains en considérant l'exigence d'efficacité économique et en consolidant la jurisprudence, tels sont les objectifs de cette réforme. Si l'Assemblée nationale en première lecture a largement respecté le travail réalisé par le Sénat, des dispositions importantes restent toutefois en navette : la définition du contrat d'adhésion ; la sanction de l'abus de l'état de dépendance dans le champ contractuel la révision judiciaire du contrat, en cas de changement de circonstances imprévisible ; les sanctions de l'exécution imparfaite du contrat ; la faculté de se libérer d'une obligation dans une monnaie étrangère ; les règles applicables aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. En deuxième lecture, la commission des lois n'est pas revenue sur les modifications apportées par l'Assemblée nationale chaque fois que cette rédaction constituait un compromis raisonnable, comme en matière en matière de nullité pour réticence dolosive. Si la commission des lois avait pour volonté de proposer des amendements de compromis, elle a, en revanche, souhaité maintenir la position déjà retenue en première lecture par le Sénat sur deux points : la révision judiciaire pour imprévision, qui porte une atteinte disproportionnée au principe de la force obligatoire du contrat et altère gravement l'image du droit français ; la question de l'application de la réforme aux contrats antérieurs.

code civil doit pouvoir refléter l'état réel du droit positif, qui a évolué sous l'oeuvre de la jurisprudence et de la doctrine depuis 1804, cette réforme est nécessaire. et Territoires votera donc en faveur de la ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

les travaux du professeur Catala ayant débuté en 2005. Comme nous avons eu l'occasion de le constater, les dispositions de cette ordonnance, bien que parfois très techniques, concernent un grand nombre de nos concitoyens, puisqu'elles modifient des pans entiers de notre code civil qui encadre les encadre les relations contractuelles et obligataires et dont l'utilité est quotidienne. Dans un premier temps, je souhaite saluer le travail du rapporteur, François Pillet, qui a permis de porter dans le débat public des questions jusque-là débattues uniquement au sein de la doctrine. Compte tenu de l'importance de ces dispositions dans la vie quotidienne des Français, il aurait été impensable que la Haute Assemblée donne son quitus sans examiner dans le détail les modifications codifiées. Je ne vais pas rappeler devant vous l'ensemble des apports de ce texte fondamental, qui ont déjà été présentés en première lecture et aujourd'hui encore par vous, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur. Sur certains sujets, ces débats ont permis de mettre en lumière l'affrontement de deux philosophies. Je pense en particulier aux dispositions relatives aux clauses abusives des contrats d'adhésion et au rôle du juge dans les relations contractuelles avec l'intégration de la théorie de l'imprévision dans le droit civil. Sur ce dernier point, et en schématisant, il s'agit de se prémunir contre certaines situations rendant inapplicable le contrat. L'article 8 du projet de loi, introduit en première lecture par le Sénat, vise à cette fin à supprimer l'introduction du régime de l'imprévision dans le code civil au motif de garantir la « liberté contractuelle L'idée de confier davantage de prérogatives au juge dans le rééquilibrage des relations contractuelles nécessitera probablement des moyens supplémentaires, ce qui n'est pas le moindre des obstacles dans le contexte budgétaire actuel. En effet, l'état de nos juridictions est tel qu'une révolution budgétaire aurait certainement plus d'impact sur l'effectivité des droits de nos concitoyens que toutes les codifications envisageables. À ce stade avancé de l'élaboration législative, il convient cependant de souligner un paradoxe. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 8 du projet de loi de modernisation et de simplification du droit du 16 février 2015. L'un de ses principaux objectifs était de réintroduire davantage de sécurité juridique dans les relations contractuelles. Des contrats ont été formés sur la base des dispositions de cette ordonnance, entrée en vigueur le 1 octobre 2016, il serait malencontreux d'instiller de l'insécurité juridique, en introduisant des modifications trop grandes au coeur de la loi de ratification d'une ordonnance, justement destinée à l'effet inverse. Sans remettre en cause le bien-fondé de la position du rapporteur sur des sujets aussi essentiels que ceux que j'évoquais à l'instant, il me paraîtrait plus raisonnable de ratifier l'ordonnance sans remettre en cause l'état du droit, d'en surveiller étroitement l'application et de proposer, le cas échéant, un retour aux dispositions antérieures, si d'importants dysfonctionnements étaient constatés par la suite. Plusieurs de mes collègues l'ont déjà souligné, cette façon de légiférer est frustrante pour les parlementaires, dont le pouvoir d'amendement se trouve limité par leur volonté pragmatique de ne pas fragiliser la situation juridique d'individus concernés par l'ordonnance. Elle est aussi gênante pour le Gouvernement, qui doit anticiper l'effet contentieux des ratifications en cas de modifications substantielles portées à l'ordonnance déjà entrée en vigueur. J'ajoute que, contrairement à une idée reçue, le recours à l'ordonnance pour d'importantes entreprises de codification n'est n'est pas sensiblement moins long que le recours à la procédure législative ordinaire. À titre de comparaison, sachez que la dernière rénovation du code pénal s'était faite en six ans, depuis son dépôt au Sénat, en 1986, jusqu'à sa promulgation en 1992, qui représente moins de temps que celui qui a été consacré à la réforme actuelle du droit des contrats et des obligations, si l'on prend en compte le temps nécessaire à l'adoption du projet de loi autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnances, déposé en 2013. Dans ce contexte, compte tenu des différentes réserves que j'ai évoquées, les membres du groupe du RDSE soutiendront les amendements du Gouvernement destinés à rétablir la version initiale du texte sur les points encore litigieux, mais cela ne nous empêchera pas d'avoir un regard bienveillant sur le texte finalement

récente à cette fonction de parlementaire, que j'évoque ce texte. Fruit d'une quinzaine d'années de travaux, riches de rapports, de contributions académiques, de réflexions, d'échanges nourris par la doctrine, les praticiens du droit et les acteurs économiques,

à deux objectifs principaux : la codification de la jurisprudence qui s'est développée depuis deux siècles et le renforcement de l'attractivité du droit français vis-à-vis des investisseurs étrangers en le clarifiant et l'adaptant aux enjeux des évolutions de l'économie mondialisée. Gagner en attractivité sans renoncer à la justice contractuelle ; s'adapter aux exigences de l'économie de marché tout en protégeant les plus faibles : tel est l'esprit de ce texte, qui introduit plusieurs innovations en ce sens. Je ne ferai qu'évoquer la définition dans le dans le code civil d'un contrat d'adhésion et la consécration de l'annulation des clauses emportant un déséquilibre significatif dans ce type de contrat, le champ volontairement élargi de la réticence dolosive,

vous l'avez souligné, ainsi que notre collègue Jacques Bigot, ces dispositions ne nuisent pas à l'attractivité du droit français, puisqu'elles n'ont qu'un impact assez limité en matière de droit des contrats internationaux. Vous avez précisé le rôle du juge, qui n'a pas vocation à refaire le contrat, mais, au contraire, à rétablir la relation telle qu'elle avait été envisagée par les parties initialement. On peut même presque considérer qu'il s'agit là d'un renforcement de la volonté des parties et d'un retour au contrat.

qui,, n'a apporté que de rares modifications au regard de l'ampleur de la réforme, qui porte sur plus de 300 articles du code civil, et qui a su, en première lecture, oeuvrer pour de véritables clarifications. C'est dans le même esprit de responsabilité que la commission des lois du Sénat, en seconde lecture, a cherché avant tout une position de compromis sur les principaux points divergents. Il en est ainsi, monsieur le rapporteur, du choix fait de ne pas définir l'abus de dépendance comme relevant uniquement du domaine économique, mais de préciser qu'il n'est pas applicable à un tiers. Comme je l'ai rappelé, le Gouvernement lui-même s'est montré à l'écoute de nos travaux, puisqu'il a réintroduit une définition du contrat d'adhésion plus proche du sens que lui avait donné le Sénat, à savoir celle d'un contrat qui « comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ». C'est une voie médiane qui a été empruntée et qui permet le compromis sur un texte équilibré

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je réitère tout d'abord mes félicitations à notre rapporteur pour son travail approfondi, ses efforts de synthèse et son choix de toucher le moins possible au droit spécifique résultant de la mise en application de l'ordonnance avant sa ratification, ce qui revient d'ailleurs à mettre le Parlement devant le fait accompli ... Constatons que ce qui devait rester exceptionnel, justifié seulement par l'urgence- je veux parler de la procédure des ordonnances -, est devenu une habitude, habitude, ce dont on ne saurait se satisfaire. Vous le savez, mon groupe est pour l'abrogation pure et simple de l'article 38 de la Constitution, qui ouvre la possibilité au Gouvernement de légiférer par ordonnances. Si seulement la révision annoncée permettait d'inscrire dans la Constitution la proposition n° 20 du président du Sénat, nous ferions un pas non négligeable vers le souhaitable. Cette proposition, je le rappelle, vise à encadrer davantage le recours aux ordonnances par deux dispositions fixer à trois mois à compter de la promulgation de la loi d'habilitation le délai dans lequel les ordonnances doivent être prises ; prévoir une ratification obligatoire des ordonnances dans un délai d'un an au maximum à partir de la promulgation de l'habilitation. Comme notre rapporteur, j'attends donc avec impatience le moment où la révision constitutionnelle viendra en débat, au Parlement ou directement devant les Français, s'ils sont consultés par référendum. Je ne doute pas que ce débat, au-delà des intentions initiales du chef de l'État d'affaiblir un peu plus le pouvoir législatif, permettra, au contraire, de donner un coup d'arrêt à la dérive consulaire du régime et à la réduction du Parlement en une chambre d'enregistrement des volontés élyséennes- mes chers collègues, Pour le reste, ces propositions de réforme du droit des contrats, largement consensuelles, n'appellent pas de longs développements de ma part. Je constaterai simplement, une fois n'est pas coutume, mon accord avec l'Assemblée nationale et le le Gouvernement sur deux points du texte qui ont fait débat ici : la suppression du terme « économique » dans la définition de la notion de dépendance, qui pouvait entraîner une interprétation trop restrictive de celle-ci l'extension du rôle du juge en cas de « changement de circonstances imprévisible » avec la possibilité qui lui est donnée, au-delà du pouvoir de mettre fin à contrat de ce fait, d'en modifier les termes. À l'inverse, la définition du contrat d'adhésion proposée par notre commission permettra de bien cerner le champ d'application de ce type de contrat, qui, dans certains cas, comme les abonnements, ne résulte pas vraiment d'une négociation entre les parties.

sans avoir précisé que notre groupe votera le texte qui nous est proposé.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, ce texte constitue un bel exemple de l'apport de la navette parlementaire et de contribution de notre assemblée à la qualité du droit, sujet essentiel pour l'attractivité économique du pays et pour le développement de nos entreprises. Vous avez reconnu, madame la garde des sceaux, qu'un dialogue fructueux s'était noué depuis le début du processus de ratification avec notre assemblée pour corriger quelques malfaçons et améliorer le dispositif. Le Sénat a réellement contribué à clarifier le texte de l'ordonnance en veillant à n'en modifier ni le sens ni l'esprit.

Il faut reconnaître qu'il s'agit là d'un texte d'une technicité juridique incontestable. Aussi, je remercie une fois encore le rapporteur François Pillet, qui m'a associée aux auditions dans le cadre de la délégation aux entreprises. À l'Assemblée nationale, en première lecture, la commission des lois et le Gouvernement se sont démarqués du Sénat sur trois points principaux. Tout d'abord, la sanction de l'exploitation abusive d'une situation de dépendance par un contractant, que le Sénat a voulu réduire à la seule situation de dépendance économique. Cette restriction, à laquelle le Gouvernement s'était opposé, priverait notre droit d'un mécanisme permettant de sanctionner les abus commis à l'encontre d'un cocontractant qui se trouve en situation de dépendance psychologique à l'égard d'un autre cocontractant. Sur ce point, la commission des lois a choisi de faire un pas vers le Gouvernement et de limiter l'état de dépendance au cocontractant. Ensuite, la sanction des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans les contrats d'adhésion, comme cela existe déjà dans les contrats de consommation, par exemple. Ce choix n'a pas été remis en cause par le Sénat, mais un débat a été ouvert sur la définition même du contrat d'adhésion, qui a été modifiée par le Sénat, puis par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ces modifications successives Enfin, la révision du contrat pour imprévision, qui permet l'adaptation du contrat dont l'exécution est rendue excessivement difficile pour l'une des parties par un changement de circonstances indépendant de la volonté des parties.

pour preuve le fait que l'amendement présenté par le Gouvernement, qui tend à préciser la définition des contrats d'adhésion en remplaçant la référence « aux conditions générales » par la notion d'« ensemble clauses non négociables », ait reçu le plein soutien de notre commission des lois. En matière de sanction des clauses abusives dans les contrats d'adhésion, nous souhaitons que nos collègues députés en viennent à reconsidérer la rédaction proposée par le Sénat dans sa cohérence avec la définition du contrat d'adhésion et l'intention du Gouvernement. Seules doivent pouvoir être réputées non écrites les clauses imposées par l'une des parties, et non pas celles qui ont été librement négociées ou, en tout cas, qui étaient négociables. Sur le paiement d'une obligation de somme d'argent pouvant se faire en monnaie étrangère,

nationale est allée encore plus loin en séance publique en prévoyant la possibilité d'utiliser une monnaie étrangère en tant que monnaie de compte pour tout contrat, dès lors que le débiteur de l'obligation conserverait la faculté de se libérer en euros. La commission des lois du Sénat propose de revenir à sa rédaction initiale et souhaite obtenir du ministère de l'économie et des finances les précisions nécessaires à un vote éclairé. C'est fait ! Sur ce point, j'attire une nouvelle fois votre attention, madame la garde des sceaux, sur les effets collatéraux d'une trop large ouverture pour la vulnérabilité des entreprises françaises, notamment au regard de l'extraterritorialité du droit américain liée au simple usage du dollar. Je crois savoir que ce sujet est déjà aujourd'hui pris en compte par M. le ministre de l'économie et des finances. sur le pouvoir de révision judiciaire du contrat à la demande de l'une des parties au cours de l'exécution du contrat et sur l'application de la théorie de l'imprévision. En première lecture, le Sénat a supprimé ce pouvoir de révision. L'Assemblée nationale l'a rétabli avec l'approbation du Gouvernement,

Compte tenu de la complexité croissante du droit économique, de la vie des entreprises, il ne nous semble pas opportun de livrer en quelque sorte les magistrats judiciaires à des situations auxquelles ils ne sont pas préparés. Cela nous apparaît également incohérent, car si le Gouvernement tient vraiment à ce rôle du juge, pourquoi ne pas en faire une norme impérative ? Cette modernisation du droit des contrats, réalisée par ordonnance, ce que nous regrettons également, à l'instar de nombre de nos collègues, continuera à faire l'objet de notre vigilance. Grâce aux contacts de terrain noués par la délégation aux entreprises du Sénat, nous saurons rapidement si d'autres malfaçons subsistent et nécessitent une nouvelle intervention réparatrice du législateur.

La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission.

un point, à la suite de la lecture récente d'un commentaire qui me paraît erroné. L'ordonnance a défini à l'article 1110 du code civil deux catégories de contrat se concevant de manière symétrique, à savoir le contrat de gré de gré et le contrat d'adhésion, qui n'étaient d'ailleurs auparavant que des catégories doctrinales. L'objectif était de pouvoir asseoir dans le droit commun des contrats un nouveau dispositif de lutte contre les clauses abusives pour les contrats d'adhésion : la logique du contrat d'adhésion, c'est une partie qui impose l'essentiel du contrat à l'autre partie, sans négociation possible, de sorte qu'il existe un risque structurel de présence de clauses abusives. Telle me semble être en tout cas la philosophie ayant inspiré l'ordonnance. Je précise que ce dispositif de lutte contre les clauses abusives est une innovation, qui a suscité d'importantes contestations, de la part de la doctrine comme des praticiens. En effet, le code civil postule la liberté contractuelle et l'égalité des parties, l'encadrement des contrats structurellement déséquilibrés étant du ressort des droits spéciaux. C'est donc bien un choix politique qui a été fait sur ce point dans l'élaboration de l'ordonnance, mais nous n'avons pas voulu nous n'avons pas voulu revenir dessus, par esprit de responsabilité. La définition du contrat d'adhésion par l'ordonnance est toutefois très critiquée, car elle utilise la notion de « conditions générales ». Je n'entre pas dans le détail, nous sommes parvenus à nous entendre avec le Gouvernement à partir de la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, qui retenait le critère de négociabilité pour distinguer le contrat de gré à gré et le contrat d'adhésion. Si elle n'est pas parfaite, la rédaction que nous nous apprêtons donc à adopter aujourd'hui me paraît aussi satisfaisante que possible. Je veux profiter de cette prise de parole pour clarifier un problème d'interprétation récurrent à propos du contrat d'adhésion, qui a été soulevé par des universitaires ou des praticiens concernant le contrat de société ou le pacte d'actionnaires. Un associé qui devient partie au contrat ultérieurement à la création de la société ou à la conclusion du pacte ne peut pas en renégocier les termes il doit y adhérer en bloc. Certains se demandent si, de ce fait, le pacte d'actionnaires ne pourrait pas être considéré comme un contrat d'adhésion, dont les clauses pourraient alors être contestées en raison d'un caractère prétendument abusif. Je veux préciser une nouvelle fois ce point, après l'avoir déjà fait par écrit dans mon rapport en première lecture, puis en deuxième lecture, car j'ai encore lu récemment un commentaire erroné sur cette question. Compte tenu des définitions que nous allons adopter, reposent sur le critère de la négociabilité des stipulations contractuelles, le contrat de gré à gré et le contrat d'adhésion seront chacun définis par les seules conditions de leur formation. Dès lors, l'adhésion ultérieure d'une nouvelle partie ne saurait en aucun cas avoir d'effet quant à la qualification d'un contrat de gré à gré, qui ne peut donc pas devenir un contrat d'adhésion du point de vue de cette nouvelle partie,

L'admission de l'imprévision dans le droit français des contrats est l'une des dispositions les plus emblématiques de l'ordonnance du 10 février 2016, dont nous débattons actuellement. L'imprévision est aujourd'hui admise dans de très nombreux droits étrangers et dans les conventions du commerce international.

Seule la révision du contrat en cas d'imprévision permet de rétablir l'économie générale du contrat telle qu'elle a été voulue par les parties, lorsque des circonstances indépendantes de leur volonté l'ont bouleversée. Conscient de l'atteinte susceptible d'être portée au principe de force obligatoire du contrat, le Gouvernement a donc strictement encadré la possibilité de révision judiciaire de ce contrat. Trois types d'encadrement apparaissent. Il faut tout d'abord un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du contrat, ce qui était raisonnablement prévisible restant ainsi à la charge des parties. Il faut ensuite que l'exécution du contrat soit devenue excessivement onéreuse pour une partie. Une augmentation du prix, par exemple, rendant l'approvisionnement plus coûteux, ne suffit pas à remettre en cause, à lui seul, le contrat. Il faut enfin que la partie lésée n'ait pas accepté dans le contrat d'assumer le risque d'un tel changement de circonstances. Les parties peuvent en effet toujours écarter toute possibilité de révision du contrat en cas d'imprévision. Vous aurez par ailleurs observé que priorité est donnée à la renégociation du contrat par les parties et à l'accord amiable. amiable. Le recours au juge ne peut s'envisager qu'en cas d'impossibilité de parvenir à un accord sur une révision amiable ou sur une résolution du contrat. L'atteinte portée à la force obligatoire du contrat et à la liberté contractuelle est d'autant plus à relativiser que l'article 1195, dans sa rédaction initialement proposée par l'ordonnance, est supplétif de volonté, c'est-à-dire que les parties sont libres, non seulement d'en écarter l'application, totalement ou partiellement, mais également d'en aménager librement les modalités, par exemple en définissant les changements de circonstances admis ou en prévoyant un processus spécifique de révision. Si j'entends bien les inquiétudes que certains d'entre vous expriment, elles me semblent excessives. En effet, je vous rappelle que les pouvoirs du juge sont strictement encadrés par les principes de procédure civile, en particulier par celui par celui selon lequel le juge ne pourra se prononcer que dans le cadre des demandes qui lui sont formulées. N'autoriser la révision judiciaire du contrat qu'en présence d'un accord des parties pour saisir le juge, comme le propose votre commission, me semble réduire considérablement l'utilité et l'effectivité du texte. Il est en effet à craindre que celui qui bénéficie du changement des circonstances ne soit que fort peu incité au dialogue, dès lors que son obstruction empêcherait toute perspective de révision judiciaire du contrat. En outre, il me semble qu'il serait regrettable que le juge, constatant que les conditions de l'imprévision sont réunies, n'ait d'autre choix que de mettre fin au contrat, avec les conséquences que cela peut parfois emporter, notamment d'un point de vue économique. par l'ordonnance pour l'article 1195, à laquelle je vous demande donc de revenir, permet au contraire à la partie lésée par un changement de circonstances imprévisibles de passer outre la mauvaise volonté de son cocontractant pour demander au juge de restaurer l'équilibre initialement envisagé par les parties. Que l'on s'entende bien, il s'agit pour le juge non pas de refaire complètement le contrat et de rechercher un équilibre objectif entre les prestations,

L'ordonnance fait entrer dans le droit français une notion toute nouvelle qui n'existait pas : la révision en cas d'imprévision. Le Sénat est d'accord ; il n'y a pas de contestation sur ce point.

Par ailleurs, si un cocontractant seul demande la résolution, le juge peut la prononcer. Nous ne changeons rien, car nous sommes d'accord. Le seul point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est l'hypothèse dans laquelle une seule partie

la responsabilité du juge peut éventuellement être engagée par la suite. C'est d'ailleurs ce que nous ont dit les magistrats que nous avons auditionnés, lesquels ne se sont pas montrés empressés à l'idée de se voir attribuer cette nouvelle mission dans le cadre de leurs fonctions judiciaires. Surtout, si le texte reste en l'état, il sera systématiquement écarté, dès lors qu'un conseil quelque peu avisé

certaines opérations internes se dénouent habituellement en devises, c'est-à-dire dans une autre monnaie que l'euro. La rédaction actuelle de cette disposition pourrait donc fragiliser de telles transactions. C'est notamment le cas dans certains secteurs comme l'aéronautique ou la pâte à bois-

Le présent amendement vise donc à compléter le texte initial pour englober ces pratiques en autorisant le paiement en devises pour des opérations entre professionnels lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis dans le secteur concerné. Il tend, par ailleurs, à insérer un texte spécifique dans le code monétaire et financier sur les instruments financiers à terme, communément appelés « produits dérivés », et sur les opérations de change au comptant. En effet, dans ces opérations, le paiement peut être exigé en devises s'il s'agit, par exemple, d'échanger une monnaie nationale contre une monnaie étrangère, alors même que l'opération n'a pas nécessairement un caractère international.

moyens de résister à certaines dérives qu'ouvre cette facilité du fait même de l'usage qu'en font les États-Unis, peut-être serait-il bon de persévérer, même si c'est dans l'erreur.

l'ensemble du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Mes chers